Si la France apparaît comme un très bon élève dans le bilan mondial des émissions de CO2, elle le doit, qu'on le veuille ou non, à sa production d'électricité d'origine nucléaire.

l'article. Enfin, le Gouvernement agit afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire la consommation d'énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à 2012. Mais force est de constater que les biocarburants sont les grands absents et les oubliés de ce projet de loi Énergie et climat. Que de rendez-vous manqués, de voeux pieux formulés dans le cadre des dernières lois de finances pour finalement détricoter à l'Assemblée nationale les votes du Sénat ! finances passent, les lois consacrées à la croissance verte et la loi d'orientation des mobilités aussi, mais la fiscalité des biocarburants n'évolue pas. Je souhaite évoquer les véhicules fonctionnant à l'essence, mais également les hybrides. Les Français ne s'y trompent pas : ils ont bien conscience qu'en utilisant notamment du bioéthanol, ils réalisent de sérieuses économies. De même, j'en viens au transport aérien pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement, les biocarburants font maintenant figure de solution incontournable. La France a un rôle primordial à jouer. De grands groupes comme des start-up françaises innovantes proposent des solutions complémentaires pour développer ce marché et contribuer au verdissement du transport aérien.

à l'horizon de 2030, contre 17 % aujourd'hui, il nous faut développer l'éolien en mer et, notamment, l'éolien flottant en Méditerranée. Cette énergie est la plus prometteuse en termes de puissance et d'acceptabilité, car les éoliennes sont positionnées-

Faut-il vous rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Commission européenne pour des infractions répétées de la France en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ?

la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. C'est ce qu'il convient de faire ; il nous faut réussir ! Comme l'indique le bilan annuel du programme scientifique international, les émissions de CO2 continuent d'augmenter dans le monde, à l'inverse des promesses faites lors de la conclusion

Les principaux pays émetteurs sont la Chine, l'Inde et les États-Unis, qui consomment de plus en plus de charbon et de pétrole. Les émissions européennes baissent très légèrement, à hauteur de 0,7 % en 2018.

force est de constater qu'il reste un formidable allié dans la lutte contre le réchauffement climatique et peut permettre la nécessaire transition. Pour information, la Suède, souvent citée en exemple, a divisé par deux ses émissions de CO2 entre 1970 et 1990,

en Pologne, le Président Macron avait promis des mesures « historiques et structurantes » en matière de transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques. À ce jour, ni la LOM ni la programmation la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, ne semblent corroborer les annonces présidentielles. Pourtant, il y a une véritable urgence à agir en matière écologique et climatique, comme l'ont réaffirmé en commission les quand bien même cette disposition législative n'a qu'une portée symbolique. On dit, dans un tel cas, que la mesure a au moins le mérite d'exister,

Je rappelle que les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines ont provoqué une augmentation de la température d'environ 0,74°C en un siècle.

Les conséquences du dérèglement climatique sont multiples et alarmantes- fonte des glaciers, montée du niveau de la mer, désertification, dégradation des systèmes agricoles, augmentation de l'activité cyclonique ... -et constituent une source de grandes souffrances et de destructions dans nos territoires et ailleurs. L'outre-mer en est la première victime ! C'est pourquoi nous attendons beaucoup de votre politique écologique et énergétique et nous

diviser par six les émissions de gaz à effet de serre, atteindre la neutralité carbone en 2050, réduire l'utilisation d'énergies fossiles de 40 % d'ici

Mais la réalité est que, aujourd'hui, les énergies renouvelables ne représentent que 36 % du mix énergétique à La Réunion, 20 % en Guadeloupe, 13 % en Nouvelle-Calédonie, 7 % en Martinique, 5 % à Mayotte Pourquoi les outre-mer sont-ils si loin du compte ? Parce que le Gouvernement n'a pas donné suffisamment de moyens pour atteindre ces objectifs ambitieux. En 2010, il a stoppé net les incitations fiscales pour les investissements dans le photovoltaïque. La filière, qui commençait à émerger, s'est effondrée. De même, entre 2012 et 2014, l'État a construit des centrales thermiques fonctionnant au diesel dans plusieurs territoires ultramarins,

qualifié de cavalier législatif, visant à attribuer à l'autorité de police la possibilité d'interdire la circulation sur les routes nationales des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit, pour des motifs liés à l'environnement, à la sécurité publique et à la sécurité routière. Je regrette que l'irrecevabilité de cet amendement ait

En effet, il recouvre des enjeux énergétiques, économiques, environnementaux et de sécurité. L'hydroélectricité représente de 12 % à 14 % de la production d'électricité nationale et 61 % de la production d'électricité d'origine renouvelable. La Commission européenne a mis la France en demeure de se mettre en conformité avec l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en procédant à la mise en concurrence des concessions hydroélectriques arrivant à échéance. Conformément aux principales dispositions désormais applicables au renouvellement des concessions hydrauliques, à la suite de l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'État a la possibilité de recourir à des partenariats public-privé pour exécuter ces contrats. Je voudrais saluer les initiatives prises par les collectivités, notamment par le département des Hautes-Alpes, qui a récemment décidé de participer, le cas échéant, au capital des SEM hydroélectriques qui pourraient être créées. J'espère que l'État sera attentif aux ambitions des territoires, qu'il accompagnera avec bienveillance la création de ces sociétés d'économie mixte qui pourraient regrouper les concessions de plusieurs barrages, par exemple celui de Serre-Ponçon. La parole

restent extrêmement élevées au regard de l'urgence des enjeux. Dans ce contexte, les moyens nécessaires devront être disponibles, mobiliser la capacité contributive de l'État en direction des particuliers aux moyens modestes n'étant pas la moindre des questions. Quelques principes d'intérêt général devraient, me semble-t-il, guider nos débats. En dépit de l'extension totale de l'économie de marché au secteur des énergies, je pense que l'énergie de première nécessité pour les particuliers relève de la notion de bien commun. tarifaire, pour ce qu'il en reste, devra être préservée, ainsi que les tarifs réglementés, qui protègent les plus modestes dans le temps long. L'ouverture des marchés de l'électricité dans l'Union européenne s'est fondée sur le principe de libre concurrence, considéré dogmatiquement comme devant conduire à un optimum bénéfique aux consommateurs, et donc sur la destruction des monopoles existants. À ma connaissance, la démonstration de la prétendue supériorité du modèle de marché n'a jamais été faite et nous avons souvent demandé au Gouvernement, sur certaines de nos travées, des évaluations de l'efficacité des marchés du point de vue des différents types de consommateurs. Elles nous ont toujours été refusées et, jusqu'à preuve du contraire, cela me conforte dans l'idée que, dans cette industrie de l'électricité fortement capitalistique, la tarification au coût marginal est, à long terme, dans l'intérêt du consommateur particulier.

autant entraver le développement et la montée en puissance des énergies renouvelables, la France ne doit pas sacrifier son entreprise nationale, EDF, dont on sait la contribution majeure, avec tous ses personnels, à la reconstruction du pays et à sa performance économique et industrielle depuis 1946. Si l'on veut que la France réussisse sa transition énergétique, EDF devra y prendre une part majeure et décisive, sans que l'ouverture du capital après la découpe annoncée dans le cadre du plan Hercule vienne enclencher un démantèlement définitif. Nous nous opposerons, le moment venu, à la financiarisation qui s'inscrit en filigrane dans le projet annoncé. L'État doit jouer un rôle majeur dans le cadre d'une stratégie industrielle assumée et discutée avec le Parlement, loin des errements que nous déplorons, en ce moment même, Alstom et d'autres grandes entreprises françaises, sacrifiées avec leur personnel.

en effet de la première source d'énergie propre et renouvelable. Ce secteur stratégique a dégagé un bénéfice net de 1,25 milliard d'euros l'année dernière. Comment accepter, dès lors, de confier les barrages à la gestion privée, guidée par des intérêts strictement marchands ? La privatisation, c'est la mort de toute politique écologiste dans ce secteur. Comment, d'une manière plus générale, coordonner une politique énergétique si elle est laissée au Il faut ajouter que ces barrages ont été financés en partie par les impôts des Français. Les investissements sont par ailleurs amortis. Enfin, il existe un risque réel de hausse des prix de l'électricité

de production d'énergie renouvelable. S'agissant de ces petites productions, il est indispensable que soient trouvés des compromis adaptés entre les enjeux de continuité écologique, souvent avancés, et les enjeux énergétiques, qui méritent d'être reconnus. Enfin, le recours à la biométhanisation à la biométhanisation présente plusieurs avantages environnementaux et économiques. Il favorise notamment le développement d'emplois locaux non délocalisables et engendre une véritable économie circulaire dans nos territoires ruraux. Cependant, la biométhanisation peut soulever peut soulever des réticences lorsqu'elle est liée à certaines formes d'élevage ou d'utilisation intensive des terres agricoles, qui nuisent à notre bilan alimentaire et écologique. C'est pourquoi je soutiens l'idée de mes collègues de mettre en place un label de « méthanisation verte

Nous comprenons maintenant autrement, et sans doute mieux qu'auparavant, le règne végétal et son interaction avec le reste du monde. Les végétaux sont ainsi passés du statut de paysage ou d'environnement, objectif et passif,

le cadre même du vivant en général. Les végétaux sont capables d'intégrer symbiotiquement leur environnement leurs messages chimiques et de communiquer avec leurs semblables, de mémoriser puis de remobiliser des informations de manière à reconfigurer ou même coloniser un sol, de mobiliser et d'aménager leur environnement sous forme d'habitat ou de niche ; c'est ainsi que naissent les forêts et les écosystèmes. Les végétaux constituent les conditions d'émergence du vivant

nous, en reconfigurant l'espace du vivant, mais aussi de ce que nous lui faisons. Les végétaux et la nature dans son ensemble seront alors des alliés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous ne devons pas les négliger, sous peine de passer à côté d'effets bénéfiques indéniables. Ainsi,

à détricoter le service public : la remise en cause des tarifs réglementés, l'ouverture du capital des entreprises énergétiques, la disparition de certains secteurs industriels où la puissance publique était présente, la privatisation des barrages hydroélectriques

ses alinéas 2 à 4 visent à inscrire parmi les principaux objectifs de politique énergétique française le développement de la cogénération. Si ce développement a bien évidemment un intérêt énergétique majeur dans certains pays, ce n'est pas le cas en France, puisque nous bénéficions déjà d'une production d'électricité faiblement émettrice de carbone. Ainsi, la cogénération ne peut pas constituer en elle-même une priorité de la politique énergétique ; nous devons plutôt nous concentrer sur la réduction des émissions de la production de chaleur, par exemple, en privilégiant des technologies qui disposent du meilleur rendement. C'est ce que nous faisons au travers du fonds chaleur. Un peu plus loin à l'article 1, un amendement adopté par la commission a mis en avant l'usage énergétique de la biomasse, en précisant les usages spécifiques de l'agriculture et de la sylviculture. Si l'usage de la biomasse à des fins énergétiques est nécessaire au regard de l'objectif de neutralité carbone, il apparaît également nécessaire de mentionner l'usage « matière » de la biomasse et de rappeler la nécessité de respecter la hiérarchie des usages. Il est donc proposé de préciser cet alinéa. de fixer des priorités pour la réduction des consommations d'énergie fossile en mettant fin en premier lieu à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. Cette rédaction est redondante avec le 3° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, qui prévoit déjà que l'objectif de réduction de consommation des énergies fossiles est modulé par énergie fossile. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa. L'article L. 100-4 du code de l'énergie a vocation à fixer des objectifs principaux, et l'ajout d'un sous-objectif en 2028 pour un objectif final en 2030 ne paraît pas opportun. Nous proposons également de supprimer cette En matière d'hydroélectricité, l'amendement adopté par la commission fixe un objectif chiffré de 27 gigawatts en 2028. Il s'agirait de la seule filière pour laquelle un tel objectif de capacité installée serait inscrit dans la loi.

consiste à aller vers une remise en concurrence des concessions échues dans le cadre du droit de la concurrence, sachant que les barrages resteraient propriété de l'État et que les concessions seraient regroupées avant remise en jeu

que nous prévoyons bien un nouveau parc éolien en mer en Bretagne- le débat public sera lancé très rapidement -, puis deux nouveaux parcs dans la zone Méditerranée, l'un en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'autre en région Occitanie. Néanmoins, il ne paraît pas souhaitable de mentionner explicitement cette filière par rapport aux autres. Les objectifs de 1 gigawatt

Ce sous-amendement a pour objet de conserver la précision rédactionnelle apportée par l'amendement du Gouvernement à l'objectif de « valorisation de la biomasse à des fins énergétiques », tout en retirant les suppressions d'objectifs envisagées.

crée des tensions avec le monde de l'élevage. La valorisation de la biomasse à des fins énergétiques doit se faire sans concurrence avec les productions alimentaires. Il faut éviter de suivre le modèle allemand : en 2014, près de 7 % de la surface agricole de l'Allemagne était consacrée à la méthanisation ; entre un quart et un tiers des surfaces de maïs cultivées dans ce pays sont dévolues à la production d'énergie.

pour les territoires, l'environnement et les agriculteurs. C'est pourquoi cet amendement vise à établir clairement qu'il convient de ne pas organiser de concurrence entre production alimentaire et production d'énergie. S'il est intéressant de valoriser la biomasse à des fins énergétiques et de développer une méthanisation raisonnée, dimensionnée à la ferme et au territoire, la laisser empiéter sur la production alimentaire serait une grave erreur. L'amendement

agricole et la production de biogaz au titre des objectifs de la politique énergétique française. Le gaz renouvelable constitue l'un des moyens de la décarbonation du secteur énergétique et des transports et de l'indépendance énergétique des territoires.

une attention spécifique est portée à la conciliation de cette production d'énergie avec l'agriculture. L'amendement

est d'inscrire dans la loi, en conformité avec la priorité donnée au développement des énergies renouvelables, la possibilité de produire de l'énergie hydroélectrique

la réflexion sur le développement de la production d'électricité à partir de l'énergie des marées. Madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, peut-on être indifférent à un process

Ce que je sais, c'est que la capacité énergétique identifiée représente l'équivalent de 15 gigawatts,

L'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable qui a l'avantage non seulement d'être décarbonée, mais aussi de permettre le maintien des réseaux. Au regard de la pertinence de cette énergie et des difficultés de développement que rencontre en particulier la petite hydroélectricité dans certaines régions,

: La parole est à M. Éric Gold. Le projet de loi reprécise la trajectoire vertueuse d'augmentation de la part d'énergies renouvelables. Il s'agit évidemment non pas d'y mettre un frein, mais de l'encadrer, car la ressource en eau n'est pas une ressource comme les autres.

227 vont à l'encontre des orientations fixées par la commission concernant le biogaz, l'hydroélectricité, l'éolien en mer, mais aussi la production simultanée de chaleur et d'électricité et la sortie des énergies fossiles. Elles constituent un signal négatif pour les professionnels de ces secteurs, qui comptent sur le soutien effectif des pouvoirs publics pour réussir la transition énergétique. En outre, dans la mesure où les objectifs fixés par la commission sont inspirés de la PPE en cours de révision -pour ce qui concerne l'hydroélectricité -ou de la dernière déclaration de politique générale du Premier ministre

à l'amendement n° 227, qui vise à supprimer l'ensemble des dispositions problématiques tout en conservant la réécriture de l'objectif de valorisation de la biomasse, qui est pertinente. pertinente. L'amendement n° 321 rectifié vise à promouvoir l'autoconsommation parmi les objectifs de la politique énergétique. Cet ajout n'est pas opportun puisque la commission a déjà prévu, au présent article, que la PPE comprenne une « stratégie pour le développement des projets de production d'énergie renouvelable » destinée à favoriser de tels projets.

est satisfait puisque les dispositions générales relatives à la biomasse introduites par le sous-amendement précité trouveront à s'appliquer au cas plus spécifique de la méthanisation.

pour atteindre 2 000 mégawatts supplémentaires entre 2016 et 2028, en réservant un quart de cette augmentation à la « petite hydroélectricité Ce chiffrage reste cohérent avec le projet de PPE, qui prévoit une cible haute de 26,7 gigawatts de capacités de production installées en 2028, ainsi qu'avec l'article 6 B du présent projet de loi, qui facilite l'augmentation de puissance des installations existantes.

certains lui reprochant de fragiliser l'élevage et de privilégier la production d'énergie au détriment de la production alimentaire. Il ne faudrait pas que certaines entreprises mobilisent l'essentiel des ressources végétales au profit de la méthanisation tant qu'il en est temps, tirons les leçons de l'expérience allemande et de ses excès. Peut-être faut-il envisager soit une charte de bonne conduite, soit un label de « méthanisation verte »- Angèle Préville avait déposé un amendement à cette fin -, soit des mesures de prévention et un régime de sanctions.

La séance est reprise. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 168 rectifié,

il serait illogique, voire contradictoire, que le développement d'une politique énergétique respectueuse de l'environnement ne respecte pas l'environnement et la société ! La formule que nous proposons permettra de mieux reconnaître les opérateurs de la croissance verte, qui visent la performance sociale et environnementale de leur activité. l'énergie, qui définit les objectifs de la commission de régulation de l'énergie, la CRE, renvoie aux deux premiers articles du code de l'énergie.

Ainsi adapté, notre cadre législatif permettra aux acteurs du secteur énergétique de mieux prendre en compte les objectifs de développement durable, les ODD, auxquels la France a souscrit en 2015 dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations unies.

prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité.

que géographique : il n'apparaît ni dans le code de l'énergie ni dans le code de l'environnement. En outre, cet amendement est doublement satisfait par les modifications apportées en commission : d'une part, la définition de la neutralité carbone mentionne les puits de carbone ; de l'autre, l'objectif relatif à la biomasse fait référence à la nécessité de préserver les sols. Les puits de carbone, tels que la forêt et la mer, sont donc pleinement pris en compte au titre des objectifs de la politique énergétique.

Le projet de loi inscrit la neutralité carbone parmi les grands objectifs de la politique énergétique : celle-ci suppose bien sûr de développer les puits naturels de carbone pour compenser les émissions résiduelles que nous ne saurons pas éradiquer.

Il est nécessaire de planifier et de préparer concrètement la sortie des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables, et de réduire la consommation d'énergie de manière générale. Avec cet amendement, nous souhaitons faire en sorte que les déclarations d'objectifs soient concrètement suivies d'effet, par le biais d'une véritable programmation en matière énergétique et de lutte contre le changement climatique.

loi permettra au Parlement de définir tous les cinq ans les objectifs et les priorités d'action des pouvoirs publics dans les domaines de l'énergie et du climat. Il est même prévu

Lienemann. Cet amendement vise à reprendre l'avis du CNTE, qui souligne l'attention particulière devant être portée à la réduction de l'empreinte carbone engendrée par la consommation de produits importés.

Ceux comportant le plus de co-bénéfices par rapport aux objectifs de développement durable prévoient un renforcement de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement d'ici à 2030. Le GIEC indique dans son rapport

et non pas seulement climatique -, il n'est plus temps de revoir les objectifs à la baisse ni d'en rester à de simples déclarations. L'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 correspond à l'engagement pris par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de Paris de 2015. le rythme de la transformation nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 est aujourd'hui insuffisant, comme le souligne le rapport du Haut Conseil pour le climat.

le souligne le Haut Conseil pour le climat, il faut renforcer les actions dès à présent. Cet amendement vise donc à réajuster et à accentuer nos objectifs en fonction d'une projection des émissions nationales prenant en compte des critères d'équité entre pays. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont en nette augmentation, plus de 2 % en 2018. Nous sommes devant un défi planétaire ; il n'est plus temps d'attendre que les autres pays agissent, chacun doit prendre sa part de responsabilités. Notre planète nous est commune, nous devons prendre les devants et faire le maximum,

Notre objectif n'est plus de diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4 car il est maintenant bien plus ambitieux : les diviser par 8 pour atteindre zéro émissions nettes en 2050. Le @gouvernementFR va le mettre dans la loi, c'est inédit ! » Ainsi

Atteindre la neutralité carbone suppose de diviser par huit les émissions de gaz à effet de serre, comme l'avait initialement indiqué le Gouvernement. Le projet de Stratégie nationale bas-carbone, ou SNBC, indique que les émissions doivent être réduites de 83 % en 2050 par rapport à 2015. Cela correspond à une réduction des émissions de de 85,8 % par rapport à 1990, c'est-à-dire à leur division par sept. Cependant, le projet de SNBC inclut des puits technologiques de carbone

d'après le scénario dit « avec mesures supplémentaires », ou AMS, sur lequel se fonde le Gouvernement, le facteur de réduction permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050 est précisément de 6,8 ou de 8, selon que l'on tient compte ou pas des nouvelles technologies. Dès lors, retenir un « facteur supérieur à 8 supérieur à 8 » apparaît très ambitieux, voire irréaliste. Rappelons que, selon le scénario du Gouvernement, il faudra déjà décarboner presque intégralement notre système énergétique et diviser par deux notre consommation énergétique d'ici à 2050 pour atteindre l'objectif de division des émissions de gaz à effet de serre par un « facteur supérieur à 6 ». C'est pourquoi il est préférable d'opter pour une hypothèse plus crédible. Les amendements n 256, 257 rectifié, 159, 188 et 159 visent à relever de 40 % à 57 % le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Or le scénario prévoit une baisse de 40 % des émissions en 2030, dans le but d'atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de modifier un objectif cohérent avec la division « par un facteur supérieur à 6 » des émissions en 2050. viser une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 17 points supérieure à celle prévue mettrait sous tension notre modèle énergétique et certains secteurs d'activité, qui n'auraient pas nécessairement le temps d'évoluer en une dizaine d'années tout au plus. Enfin, l'amendement n° fixer des objectifs de réduction de l'« empreinte carbone de la France ». L'empreinte carbone est une notion intéressante, qui offre une vision d'ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées par la consommation nationale, puisqu'elle intègre les importations. Pour autant, cet indicateur pose des difficultés

pour éviter des effets juridiques non anticipés sur les documents de planification et le soutien aux projets publics. Il n'apparaît donc pas judicieux d'intégrer parmi les objectifs de la politique énergétique un outil encore mal défini. En conclusion, la commission est défavorable à l'ensemble de ces amendements.

L'objectif de neutralité carbone en 2050 que le Gouvernement a retenu dans ses projets de Stratégie nationale bas-carbone a été validé par le Haut Conseil pour le climat. Ce dernier a en effet considéré que cette trajectoire compatible avec un objectif d'augmentation des températures limitée à 1,5 C, que l'ambition est satisfaisante et que les sous-objectifs sont cohérents par rapport à l'ambition générale. La trajectoire sous-jacente à la SNBC et à la PPE respecte ainsi l'objectif intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et aboutit à une réduction prévisionnelle légèrement supérieure aux 40 % visés. Elle repose sur des mesures déjà très ambitieuses et fait de la France un pays leader en matière d'objectifs. En ce qui concerne la réduction de l'empreinte carbone elle-même, le Gouvernement souscrit pleinement à l'objectif de sa réduction pour couvrir aussi le carbone importé.

Néanmoins, la mesure de l'empreinte carbone est soumise à de nombreuses incertitudes méthodologiques. Elle dépend du contenu carbone des moyens de production des autres pays. Pour ces raisons, la réduction de l'empreinte carbone ne peut pas se piloter comme la réduction des émissions du périmètre sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°

considérant que les calculs ont été faits sur une réduction compatible avec un facteur supérieur à six, mais pas avec un facteur supérieur à huit : nous ne sommes pas en mesure d'avoir cette ambition. Par ailleurs, c'est un facteur de l'ordre de six qui permettra d'atteindre notre objectif global.

M. Jean-Pierre Decool. L'exclusion de toute compensation par des crédits internationaux dans la définition de la neutralité carbone a été introduite par la voie d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale. Elle n'a fait l'objet d'aucune étude impact ni d'aucun véritable débat. Or la définition de la neutralité carbone dans la loi française ne doit pas donner l'impression d'empêcher les entreprises et les territoires d'agir à l'international et de développer une coopération Nord-Sud utile pour les populations locales, notamment en Afrique, en utilisant la flexibilité offerte par les crédits carbone internationaux. Cette définition doit être cohérente avec l'accord de Paris, dont l'article 6 prévoit explicitement la coopération internationale, et en particulier l'utilisation de crédits carbone internationaux comme moyen pour réussir à atteindre son objectif. Plusieurs États européens, dont la Norvège et le Royaume-Uni, qui visent un objectif de neutralité carbone à court ou moyen terme, semblent s'engager dans la voie de la compensation par des crédits internationaux. Il ne faudrait pas que l'interdiction française pénalise nos entreprises et la mise en oeuvre de projets de coopération internationale. la neutralité carbone semble porter sur l'inventaire national, et non sur le bilan carbone des entreprises, il est important que le Gouvernement le confirme publiquement, afin de rassurer les entreprises et de dissiper les doutes.

de la prise en compte des crédits internationaux de compensation carbone dans la définition de la neutralité carbone a été introduite à l'Assemblée nationale. Cette exclusion n'a pas été supprimée par la commission aux fins, d'une part, de rechercher un consensus sur les grands enjeux climatiques, et, d'autre part, de porter à un haut degré d'exigence les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La neutralité carbone étant un objectif mais ne produisant pas d'effets juridiques, elle laisse totalement inchangés les mécanismes de compensation carbone issus du protocole de Kyoto, qui conservent par ailleurs toute leur utilité pour accompagner les pays émergents dans leur transition énergétique.

Cet objectif n'exclut évidemment pas ceux de solidarité climatique et d'aide au développement fixés dans le cadre de l'accord de Paris. La France s'implique très fortement, notamment l'Agence française de développement. Enfin, cet objectif n'est pas applicable aux entreprises. Nous parlons ici du budget carbone français

Il s'agit de préciser les objectifs de réduction de consommation de l'énergie finale dans le temps, de 2023 à 2030, en relevant à 22 % l'objectif de réduction fixé pour 2030, comme le propose le réseau Action Climat. Le rythme actuel de réduction de la consommation énergétique finale est insuffisant. En effet, une analyse des trajectoires pour atteindre une réduction de 50 % de la consommation d'énergie en 2050 indique que la baisse devrait être au moins de 22 Il est donc nécessaire de réviser la trajectoire et d'engager un effort sans précédent en faveur des économies d'énergie, qui doivent être la priorité absolue de la politique énergétique. La recommandation émise le 18 juin par la Commission européenne précise d'ailleurs que la France doit détailler les politiques et mesures mises en place afin d'atteindre les objectifs de réduction de sa consommation énergétique finale.

s'agit d'avancer de manière progressive et régulière. L'analyse des trajectoires, pour atteindre une baisse de 50 % en 2050, indique un point de passage en 2030 à 22

de 50 % en 2050. Une telle ambition impose anticipation et adaptation des modes de consommation d'énergie de l'ensemble des secteurs, afin de répartir les efforts à effectuer dans le temps. C'est dans ce cadre que le Conseil supérieur de l'énergie s'est prononcé en faveur de l'établissement de jalons intermédiaires, en vue de tracer clairement la trajectoire de réduction de nos consommations d'énergie d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050.

supplémentaires, les premières baisses de consommation d'énergie, par exemple les émulations écologiques, étant les plus faciles à obtenir. Ce rehaussement de l'objectif peut également apporter un gain de pouvoir d'achat à court terme, en réduisant l'impact de la hausse du prix des énergies sur les budgets des ménages,

388 rectifié visent à fixer des jalons intermédiaires pour garantir l'atteinte de l'objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique finale d'ici à 2050.

Par ailleurs, l'article 1 fixe déjà un objectif intermédiaire, adopté par l'Assemblée nationale et conservé par la commission, prévoyant une réduction de 7 % de la consommation énergétique finale en 2023. Je pense que nous devons nous garder de fixer des objectifs trop ambitieux pour pouvoir être atteints au regard des scénarios de référence et de multiplier les jalons : cela nuit à la lisibilité et à l'appropriation des objectifs.

de poser des jalons complémentaires d'ici à 2030. Par ailleurs, le projet de loi fixe un objectif de réduction de 20 % de la consommation énergétique en 2030. Cet objectif est en réalité déjà extrêmement ambitieux

Je suis conscient que l'effort envisagé devra sans doute être ajusté d'ici à la conclusion de nos travaux, mais je suis convaincu de la nécessité d'inscrire dès à présent l'objectif dans le projet de loi. Je constate également que cet objectif est cohérent avec l'amendement

AMS », servant de base à la révision des objectifs du projet de loi, de la PPE et de la Stratégie nationale bas-carbone, et nuirait à la cohérence d'ensemble de la trajectoire en faveur de la transition énergétique. Il va d'ailleurs être difficile de tenir cette trajectoire, compte tenu du retard annoncé dans la mise en service la mise en service de l'EPR de Flamanville. En deuxième lieu, un arrêt précipité du recours à l'énergie nucléaire n'est pas compatible avec nos engagements climatiques. faute d'un développement suffisant des énergies renouvelables et des capacités de stockage de l'électricité, la réduction de la production d'énergie nucléaire pourrait entraîner un report de la consommation vers les énergies fossiles, et une augmentation des émissions de gaz à effet Dans ce contexte, une dégradation de la sécurité d'approvisionnement, du coût de la fourniture d'électricité et de la balance des paiements est à prévoir.

sans pour autant déterminer les moyens de les atteindre, en totale incohérence avec l'urgence écologique et climatique. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la rénovation des bâtiments. Ce secteur, qui représente 44 % de l'énergie consommée en France, France, a pourtant fait l'objet d'un plan, présenté il y a bientôt deux ans : 14 milliards d'euros devaient être consacrés, sur le quinquennat, au financement de la rénovation de 500 000 logements par an,

L'article L. 100-4 du code de l'énergie fixe comme objectif très ambitieux la rénovation de l'ensemble du parc immobilier selon les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées à l'horizon 2050, une politique de rénovation thermique des logements ciblant prioritairement les ménages aux revenus modestes. Le présent amendement vise à retranscrire en tant qu'objectif intermédiaire l'engagement pris par le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron de rénover un million de logements mal isolés d'ici à 2022, en accordant la priorité aux ménages les plus modestes. Nous espérons que le projet de loi de finances donnera

Tout d'abord, prévoir que la politique de rénovation énergétique concernera prioritairement- et non plus majoritairement -les ménages modestes reviendrait à réduire les ambitions de cette politique à l'égard de ces derniers.

Enfin, sur l'initiative de la commission, le champ de la loi quinquennale instituée par l'article 1 A a été complété pour tenir compte de la nécessité de fixer des objectifs en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Le législateur aura donc l'occasion de redéfinir

les enjeux énergétiques liés aux transports pourront tout à fait être abordés tant dans le cadre du volet de la PPE institué par le présent article, portant sur l'identification des usages pour lesquels la réduction de la consommation d'énergie est prioritaire,

Engager la transition vers une mobilité propre est au coeur du projet de loi d'orientation des mobilités et des objectifs du Gouvernement. Cette transition ne peut s'envisager qu'au travers du report modal vers le rail. Le projet de loi d'orientation des mobilités inscrit pour la première fois dans notre droit l'objectif, fixé dans le plan Climat, d'atteindre la neutralité carbone pour les transports terrestres d'ici à 2050. Il s'agit de réorienter les investissements en faveur de transports propres au quotidien. Le texte prévoit ainsi une hausse de 40 % des investissements de l'État dans le transport durant le quinquennat, avec une réorientation claire en faveur des transports du quotidien trois quarts des investissements du quinquennat seront dédiés au ferroviaire. Le projet de loi d'orientation des mobilités prévoit également de grandes avancées pour la mobilité électrique. L'objectif est de multiplier par cinq les points de recharge pour les véhicules électriques d'ici à 2022, avec l'équipement obligatoire en bornes pour les parkings de plus de dix places des bâtiments neufs.

à l'horizon 2030. Elle a ainsi d'abord étudié le potentiel d'énergies renouvelables disponibles et mobilisables dans ces trois territoires. Selon les estimations de l'Ademe, la production annuelle d'électricité à partir d'énergies renouvelables représenterait entre 35 % et 53 % de la production totale en 2030 pour la Guadeloupe et La Réunion. En Martinique, les gisements renouvelables pilotables étant moins importants, cette part serait comprise entre 58 % et 73 % en 2030. En clair, atteindre l'autonomie énergétique est impossible, sauf à fournir un effort supplémentaire de maîtrise de la demande d'énergie, couplé à une accélération du déploiement des énergies renouvelables.

de réaffirmer ici que l'État se doit de donner aux territoires ultramarins l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de cette obligation légale. Quel

il est préférable de conserver une date suffisamment souple pour qu'elle puisse être tenue. Par ailleurs, la formulation de cet objectif afférent aux départements d'outre-mer n'est pas seule à comporter la notion d'« horizon puisque le droit existant fixe un objectif de rénovation énergétique « à horizon 2030 » et le présent article l'atteinte de la neutralité carbone « à horizon 2050 ». L'avis est défavorable.

à figer le droit, alors que les technologies évoluent très rapidement dans ce domaine. Enfin, relevons que la transition énergétique, dans les départements d'outre-mer, ne passe pas uniquement par l'énergie solaire, comme pourrait le laisser croire cet amendement, mais aussi par l'hydroélectricité, la géothermie ou la biomasse.